La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. En conséquence, nous pourrions retirer de l'ordre du jour, en accord avec le Gouvernement, les conclusions de la commission mixte paritaire ou l'examen en nouvelle lecture de ce projet de loi,

suspension de séance. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental

nom du peuple français, lequel n'intervient jamais dans la justice, qui est rendue par des magistrats professionnels, sélectionnés parce qu'ils ont la formation et les compétences pour rendre des décisions de justice. Le tirage au sort permet de réintroduire les citoyens français dans le processus de justice, qui se déroule en leur nom. Il n'en va pas de même s'agissant de la représentation démocratique en France.

mais ce sont aussi les élus ; les élus sont des citoyens choisis parmi les autres. Alors, s'il est compréhensible que le peuple français soit réintroduit dans la justice rendue en son nom, il

Je finirai quand même sur un accord, monsieur le garde des sceaux, puisque je crois que nous tenons tous les deux autant à ce que les jurys d'assises continuent à être tirés au sort. Je suis saisie de six

De la même façon, je rappelle que le tirage au sort, qui ne doit pas être confondu avec une quelconque loterie, est un processus, un outil déjà expérimenté et utilisé, pratiquement dans les mêmes conditions que celles que nous proposons aujourd'hui, dans de nombreuses organisations, collectivités ou autres, en France ou à l'étranger. La position de la commission des lois nous apparaît ici un peu en décalage avec les attentes de la société. Si nous n'avions rien à redire, si nous pensions que tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si la démocratie était vivante, si les élus l'étaient avec 80 % de participation, peut-être pourrais-je partager votre opinion, madame la rapporteure, mais tel n'est pas le cas. En tant qu'élu et citoyen, je me dois d'essayer de trouver des outils pour faire en sorte que cette démocratie, nécessaire dans le contexte économique, social, environnemental où nous nous trouvons, puisse être revitalisée. Le tirage au sort est un de ces outils. Pour autant, il ne délégitime absolument pas la démocratie représentative. Il vient compléter, et non pas en concurrencer, la consultation de la société civile organisée. La Convention citoyenne pour le climat a montré l'intérêt de ces procédures. Des citoyens de tous milieux sociaux, et notamment issus des couches les plus modestes de la société, qui ne sont pas forcément inclus aujourd'hui dans les processus

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 tel qu'il avait été voté par l'Assemblée nationale.

Nous sommes favorables à la mise en oeuvre d'une disposition qui permette au Conseil économique, social et environnemental de faire appel à des consultations citoyennes, avec des personnes tirées au sort,

souhaitons préciser que le périmètre du public doit être représentatif de la composition de la population française du point de vue du sexe, de l'âge et des catégories socioprofessionnelles. Deuxièmement, nous prévoyons que les résultats d'une consultation feront l'objet d'un débat devant le Parlement, lorsque la consultation aura été demandée par le Premier ministre, ou devant la chambre qui aura sollicité cette consultation. concernant les résultats de la consultation, leur publication devra être faite dans un format ouvert afin de favoriser l'analyse des données. Nous considérons que la révolution numérique a violemment percuté le fonctionnement de la vie politique et de la démocratie représentative. Nous pouvons

La situation actuelle nous donne d'autres facilités pour travailler, mais pose aussi de nouvelles exigences. De même, les partis politiques ne fonctionnent plus de la même manière ni avec la même discipline d'expression. d'expression. Nous constatons ce besoin de trouver de nouvelles formes de mobilisation citoyenne, de nouvelles formes d'échanges continus entre les représentants du peuple et l'ensemble de la société. Sans ces nouveaux modes d'expression, la démocratie se perd ; elle devient consumériste : on prend quelqu'un et puis, après cinq ans, on le lâche, alors que la citoyenneté est un exercice de tous les jours, avec des échanges. Nous considérons que cette méthode peut permettre

C'est pour nous une disposition centrale de ce projet de loi. Il s'agit en réalité de permettre au CESE de procéder à des consultations publiques, y compris en ayant recours au tirage au sort, pour l'exercice de ses missions. À ce propos, madame la rapporteure, j'ai entendu le distinguo que vous faites entre le tirage au sort des jurés d'assises et ce tirage au sort. Vous avez raison, mais je veux juste dire que le tirage au sort en tant que le tirage au sort en tant que tel existe déjà dans notre droit et qu'intrinsèquement il ne peut pas effrayer. D'ailleurs, dans mon discours, j'ai mentionné les grandes démocraties qui utilisaient déjà cette voie. Les Français, nous le savons, réclament de plus en plus de démocratie participative. Les députés ont d'ailleurs renforcé les garanties entourant ces consultations afin de légitimer cette procédure. nous avons eu récemment la preuve de la capacité du CESE à mener à bien de telles consultations, avec l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat, qui est, disons-le, un véritable succès démocratique. Telles sont les raisons pour lesquelles

Il convient avant tout de s'accorder sur ce qui fait l'objet de nos discussions. En commission, Mme la rapporteure avait formulé l'inquiétude que l'inscription du tirage au sort dans la loi organique ne fragilise les fondements de notre démocratie. Mais que prévoit l'article que nous voulons rétablir ? La faculté, et je dis bien la faculté, pour le CESE d'enrichir ses travaux en désignant pour ses consultations publiques des personnes tirées au sort. C'est une faculté, j'y insiste, parmi d'autres modalités. Il n'est donc pas question ici de substituer des membres tirés au sort aux représentants de la société civile organisée, qui composent le CESE. Il n'est pas non plus question, puisque le caractère consultatif est bien précisé, de substituer le tirage au sort à la légitimité de l'élection, qui fonde notre démocratie représentative et qui, seule, peut asseoir, par le mandat, la décision souveraine. Une fois les choses clarifiées, il devrait être possible de dépasser l'opposition sèche et concurrente entre représentation et participation. L'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne dispose-t-il pas lui-même que « la loi est l'expression de la volonté générale », et que « tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, Au-delà du procédé, c'est la question fondamentale du processus qu'il faut poser. Les garanties d'égalité, de transparence et d'impartialité que nous proposons de rétablir apparaissent de nature à favoriser la pertinence et la qualité de la participation citoyenne.

mes chers collègues, je n'imagine pas que le Sénat, l'assemblée que nous formons, inscrive dans un projet de loi organique, dont l'une des caractéristiques est qu'il découle directement de la Constitution, la convention citoyenne et le tirage au sort,

les différents amendements ont un objet commun : rétablir la possibilité d'associer les citoyens tirés au sort aux travaux du CESE.

collègues, je vous trouve parfois bien timides au regard du faible poids de notre Parlement dans les institutions françaises ! Mais c'est un autre sujet. En quoi la démocratie participative renforce-t-elle la démocratie représentative ? Voilà la question centrale. Quelles formes peut-elle prendre ?

des corps intermédiaires. Nous ne sommes pas de ceux-là ; nous pensons qu'il est nécessaire d'organiser une respiration entre ces structures et d'autres formes d'expression du peuple. Or une convention citoyenne tirée au sort n'est pas la juxtaposition d'individus isolés, mais la collaboration de ces individus, qui confrontent publiquement leurs points de vue pour mieux expliciter les enjeux ; ils font eux-mêmes, entre eux, des arbitrages qui ne sont en aucun cas des décisions publiques, mais expliquent une étape qui se construit autour de propositions.

Aucun échantillon de cent cinquante personnes ne peut être représentatif de toute une société ! D'ailleurs, si l'on faisait un sondage sur la base d'un tel échantillon, la Commission des sondages le disqualifierait immédiatement et ce serait un scandale public de le publier. Troisièmement, l'autorécusation de centaines de personnes tirées au sort introduit dans la composition de cette prétendue convention citoyenne des biais considérables, qui empêchent de de la considérer comme représentative : c'est une supercherie ! Enfin, le choix des personnes qualifiées censées éclairer ces individus constitue un autre biais tout à fait manipulateur. Pire, les pouvoirs que le Président de la République leur a conférés par ses propos- la parole d'un Président, c'est de l'action ! -sont une négation des responsabilités du Parlement, qui seul a des comptes à rendre, comme nous l'a justement expliqué Mme le rapporteur, en rappelant le principe de responsabilité devant les Français qui caractérise notre relation avec nos concitoyens.

les votes extrêmes, l'abstentionnisme qui croît depuis des décennies, une génération qui, quand on l'interroge sur la démocratie, considère que le vote n'est pas la meilleure modalité de représentation des gens, et des problèmes collectifs qui se règlent non

il y a une méprise initiale sur le sens donné à l'expression « issue de personnes tirées au sort ». Ces personnes n'ont ni plus ni moins de légitimité que les autres.

cela n'est pas transposable au tirage au sort. Je ne nie pas que la démocratie représentative soit malade. D'une certaine façon, elle est malade depuis qu'elle existe.

En effet, nous considérons que cette procédure ne permet pas au CESE de remplir pleinement ses missions, à savoir un éclairage des politiques publiques et un dialogue apaisé et constructif entre les différentes composantes de la société.

Le risque d'affaiblissement du CESE par la procédure simplifiée a été identifié par le Conseil d'État, qui, dans son avis, considère que, si la procédure simplifiée permet d'accélérer l'adoption des avis du CESE, il convient de veiller à conserver un rôle essentiel à son assemblée plénière, plénière, notamment eu égard au renforcement de l'institution souhaité par le Gouvernement. De plus, l'expérimentation de cette procédure au cours du précédent mandat n'a pas suscité l'adhésion unanime des conseillers. Nous comprenons l'intérêt d'une réactivité du CESE pour coller à l'actualité politique, mais cette procédure simplifiée ne nous paraît pas la solution. D'ailleurs, on peut on peut aussi s'interroger sur l'accélération de la procédure législative et ses conséquences sur la qualité de la démocratie et du débat public : cette accélération n'est pas propice au dialogue avec la société civile, pourtant source de propositions et d'éclairages. Elle rend au contraire plus complexe la construction de compromis entre les différents groupes politiques. Vouloir embarquer le CESE dans cette accélération nous paraît plus que questionnable.

force de la décision publique ! Par conséquent, même si je peux comprendre que les garde-fous qui ont été prévus par la commission améliorent l'idée de passer en force n'importe comment, culturellement, on se trompe de choix. Ce n'est pas cela qui rend la démocratie et l'action efficaces, c'est l'inverse

sur l'écriture de la loi afin qu'elle fût la meilleure possible. J'observe que, avec le système dans lequel nous sommes maintenant

Ce système est déplorable pour la qualité de la loi. Toute phrase, tout mot de la loi s'applique à tous les Français, quels qu'ils soient, et s'applique souvent pour très longtemps. Les sénateurs et les députés

ou entendez-vous revenir à la lettre et à l'esprit de la Constitution ? Faites moins de lois, mais laissez-nous les faire les meilleures possible en appliquant la procédure normale et en donnant aussi au CESE le temps de bien faire son travail.

L'article 6 est une disposition phare de notre projet de loi. Il répond à l'objectif du Gouvernement de revaloriser le CESE et de lui donner plus de visibilité. Il constitue également une véritable simplification de la procédure d'élaboration Il s'agit plus précisément de donner un effet substitutif à la saisine pour avis du CESE d'un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social, environnemental, par rapport à un certain nombre d'autres consultations. Nous le savons tous, et ce phénomène est décrié depuis des années, nous n'avons cessé de créer de multiples organismes consultatifs, souvent peu connus, qui n'ont fait que complexifier et ralentir le processus d'élaboration des lois, ces organismes concurrençant souvent le CESE dans son champ d'expertise. Vous craignez que les études d'impact ne soient appauvries par l'abaissement du nombre de consultations, mais ce constat me semble tout à fait infondé et même contradictoire avec celui qui est également fait de la grande qualité des avis du CESE. Or cette qualité s'explique notamment par la diversité de compétences que présentent les membres du CESE. Je rappelle que la loi organique relative à la présentation des projets de loi loi prévoit que les rapports du CESE doivent être analysés dans l'étude d'impact. Enfin, c'est un dispositif équilibré qui vous est proposé. Cette substitution n'est en effet possible que sous un certain nombre de réserves et d'exceptions. Il a été choisi de conserver les consultations de collectivités territoriales, des instances nationales dans lesquelles elles sont représentées ou encore des autorités administratives indépendantes. Comme a pu le souligner le Conseil d'État dans son avis du 25 juin 2020, il s'agit donc d'une simplification bienvenue et de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE.

supprimé par la commission des lois. En effet, cette simplification est de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE sur les projets de loi entrant dans son champ de compétence et contribue à en faire le « carrefour des consultations publiques Il ne s'agit pas de sous-estimer l'intérêt des consultations préalables. C'est pourquoi des exceptions ont été prévues et étendues au cours de la navette. N'entrent ainsi pas dans le champ de la dispense de consultation les consultations des collectivités territoriales, des outre-mer et des instances de dialogue entre les collectivités territoriales et l'État, les consultations des autorités administratives ou publiques indépendantes ou encore les concertations préalables prévues par le droit du travail. Par ailleurs, je tiens à le souligner, la dispense de consultation que cet amendement tend à rétablir

que le CESE pourra être consulté si le Gouvernement le décide. Dans ce cas, l'avis des autres organismes consultatifs ne sera pas requis, l'avis du CESE s'y substituera, sauf dans un certain nombre de cas qui sont également énumérés dans ce texte. Les avis consultatifs des autres organismes seront alors requis et le CESE ne pourra pas s'y substituer. Cela signifie, d'une part, que l'on ne supprime aucun organisme-

En réalité, nous avons bien du mal à connaître le périmètre de cet article. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il n'introduit aucune simplification dans le droit existant. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable

cas ? Nous aurions pu trouver une voie médiane : d'une part, ne pas obliger le Gouvernement à ne pas procéder à des consultations, d'autre part, ajouter à la liste des exceptions toutes les structures qui ne sont pas représentées au Conseil économique, social et environnemental.

peine à trouver sa place- c'est une litote ... En dépit de ses réformes successives, il n'a malheureusement pas été en mesure de faire la preuve de son utilité et de répondre à sa mission fondamentale. Aussi, il convient de porter sa composition actuelle à ...

pour recevoir un nouveau musée consacré aux travaux publics. Il pourrait ainsi donner lieu à une réflexion approfondie sur une nouvelle destination de cet édifice emblématique de toutes les innovations architecturales et techniques introduites par Auguste Perret et être le lieu de culture et de prestige d'une activité culturelle ou sociale appropriée et identifiée cette fois

Monsieur le ministre, je vous donne l'occasion de ne pas faire d'acharnement thérapeutique sur une institution qui est en sédation profonde et continue depuis un certain nombre d'années. au passage de faire plaisir à votre collègue Roselyne Bachelot, qui sera très contente de trouver une utilisation cette fois utile à un lieu d'exception.

régulièrement, nous nous posons la question de son utilité réelle au regard de la mission qui lui est confiée. Nous l'avons rappelé, cette instance de dialogue social ne réduit pas les conflits sociaux dans notre pays, même si le dialogue se crée au sein de l'instance. Je rappelle qu'elle s'autosaisit sur 80 % de ses rapports, ce qui signifie bien que son rôle consultatif n'est pas appréhendé par les pouvoirs publics. Pourquoi ?

Les projets de loi arrivent devant le Parlement à une vitesse telle que nous avons parfois à peine le temps de rédiger nos rapports et de mener nos auditions. Par conséquent, comment consulter de surcroît une autre assemblée

Nous avons toujours plaidé pour le bicamérisme et nous pensons utile d'avoir un organisme consultatif qui éclaire la décision publique et qui, en coeur de cible, mobilise les partenaires sociaux. C'est en cela que nous avons toujours soutenu le CESE. Pourquoi le CESE semble-t-il impuissant ou mal entendu ? Est-ce sa faute ou est-ce la manière dont les pouvoirs publics, le Parlement, le Gouvernement

-pour des embauches dans les hôpitaux, un moratoire sur toutes les fermetures de cliniques et de lits et, en même temps, l'amélioration du rôle des soignants dans la prise de décision de l'hôpital public,

de vote. Je reconnais là l'humour de François Bonhomme. Après tout, à un moment, on a bien supprimé les crédits affectés au bourreau pour faire beaucoup plus que le bourreau ... En la matière, je ne souscris pas à la démonstration de Mme Lienemann. Si, en 2008, je me suis opposé à ce que l'on réduise le rôle du CESE, c'est que je considérais que, par rapport aux deux chambres, c'était justement l'organe citoyen

le prévoyait l'article 7 du projet de loi organique dans la version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, et en revenir à la répartition de ces membres au sein des quatre catégories.

Au regard de la nécessité d'assurer une plus grande représentativité de la société civile, la suppression de la catégorie des personnalités qualifiées, ainsi que la commission des lois en a convenu, s'est imposée. cette catégorie ne représentant que 17 % des membres du CESE, sa suppression n'est pas suffisante à elle seule pour répondre à l'objectif d'une réduction sensible

en proportion du nouveau nombre de membres du CESE, une augmentation, certes légère, mais réelle de leur représentation. Le nombre de cent

Ce rééquilibrage vise à poursuivre la logique induite par la réforme du 28 juin 2010 ayant amené à introduire dans cette enceinte des représentants de la vie sociale, territoriale et associative, d'un côté, et de la protection de l'environnement, de l'autre. Pour des motifs historiques et chronologiques, ces deux ensembles ne disposent pas des mêmes effectifs que les pôles représentatifs du dialogue social et du monde économique. Or les enjeux climatiques et la dégradation de la biodiversité sont de plus en plus prégnants et font l'objet d'un consensus scientifique, ce qui justifie la mobilisation d'une robuste expertise environnementale au sein du CESE.

Cet amendement vise à garantir la désignation d'un représentant de la société civile de chacune des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et leur répartition au sein de l'ensemble des pôles du Conseil économique social et environnemental. en effet de tenir compte de l'éclatement géographique de ces territoires. L'absence d'une représentation territoriale des outre-mer pourrait être considérée comme une exclusion de fait d'une partie de la société civile ultramarine.

Les caractéristiques et contraintes des outre-mer les placent du reste bien souvent aux avant-postes des problématiques sur lesquelles le CESE sera amené à se prononcer. L'environnement est un exemple emblématique, alors que 80 % de la biodiversité française se trouve dans les territoires ultramarins, dont on a coutume de dire qu'ils sont les sentinelles des changements climatiques. Dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, les initiatives de la société civile sont particulièrement dynamiques. Il conviendrait de ne pas priver le CESE de tels apports.

Mme Victoire Jasmin. Lors de son intervention en juillet 2017 en conclusion de la conférence des territoires, le Président de la République rappelait les particularités des outre-mer et soulignait : « les outre-mer sont confrontés souvent au cumul de nombre de difficultés

À travers cette diversité de situations, je veux manifester ainsi que ces grandes transitions que nous avons à vivre imposent à l'État non plus de garantir l'égalité parfaite- elle est impossible -, l'uniformité rêvée- elle peut se transformer en cauchemar -, mais bien plutôt de tenir son rôle et d'assurer une égalité des possibles et des chances et de permettre à chacun des territoires, compte tenu de ses contraintes de départ, de réussir les transitions qui sont à l'oeuvre et font le monde contemporain dans lequel nous avons à évoluer. » Cette citation d'Emmanuel Macron fait partie des éléments à l'origine de cet amendement.

qui ne sauraient justifier une représentation globale sans faire perdre au Conseil la richesse née de leur diversité. Pour cette raison, il semble indispensable que le projet de loi prévoie, au sein du troisième pôle, un représentant de la société civile pour chacun des territoires ultramarins.

au détriment des trois autres pôles. Un équilibre ayant été trouvé dans la composition du CESE, je ne pense pas qu'il nous appartienne de le modifier aujourd'hui. J'émets donc également un avis défavorable

l'amendement n° 25 rectifié, qui vise à réserver le pôle environnemental aux organismes ayant pour objet principal la protection de la nature et de l'environnement,

de l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par

Ce comité, composé de députés, de sénateurs, de membres du CESE, d'un membre du Conseil d'État et d'un magistrat de la Cour des comptes garantira un regard extérieur et une transparence dans les évolutions de la composition du CESE. CESE. Il permettra l'adaptation de la composition du CESE en fonction de l'évolution de la société, sans qu'il soit nécessaire de modifier systématiquement la loi organique.

combien de postes seront-ils réservés aux coopératives, aux mutuelles ? Comment va s'établir le rapport de force entre les différents champs des activités économiques prévues et des entreprises ?

tout à fait inopportun et nous l'avons supprimé en commission. En revanche, nous avons indiqué que le Gouvernement, qui procédera à ce travail, aura l'obligation de publier les critères mis en oeuvre pour choisir les différents représentants de la société civile organisée.

Mes chers collègues, vous le comprendrez aisément, il s'agit d'un amendement d'appel visant à réaffirmer, d'une part, le rôle des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales et, d'autre part, à souligner l'importance d'une représentation juste et équilibrée des outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental. Ce texte prévoit en effet, dans son état actuel, la disparition du groupe et de la délégation à l'outre-mer créés à l'origine pour prendre davantage en considération les préoccupations, les richesses et les spécificités de ces territoires. L'amendement déposé par le groupe RDPI, ainsi que ceux défendus par mes collègues socialistes tendant à offrir des garanties quant à la représentation des outre-mer au sein du CESE nous ont permis d'en débattre à l'instant, nous en sommes ravis. Je serai donc bref et témoignerai simplement de l'inquiétude que cette réforme suscite dans les outre-mer. Si le CESE n'a pas vocation à représenter les territoires, sa légitimité et sa crédibilité ne peuvent se faire sans eux.

des assemblées parlementaires. Nous savons tous, au Sénat, combien la délégation sénatoriale à l'outre-mer est essentielle et utile pour enrichir les travaux de notre belle assemblée. Aussi, cet amendement vise à donner un fondement législatif aux délégations du CESE. Le Conseil économique, social et environnemental dispose aujourd'hui de trois délégations : la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, la délégation à l'outre-mer et la délégation à l'évaluation des politiques publiques et à la prospective. Au regard des nouvelles missions confiées au CESE, notamment le recours à la procédure simplifiée, celui-ci ne peut faire l'économie d'organes de réflexion, d'information et d'expertise sur ces sujets transversaux. Première et plus ancienne délégation aux outre-mer parmi celles existant au sein des trois assemblées constitutionnelles, car elle a été créée en mai 2010, la délégation à l'outre-mer joue un rôle particulièrement important au Conseil économique, social et environnemental. le Président de la République a déclaré l'égalité entre les hommes et les femmes grande cause nationale du quinquennat, même si les moyens mis à disposition pour cette grande cause nationale demeurent insuffisants. Pour autant, il me paraît inconcevable qu'une telle délégation disparaisse alors qu'elle contribue à construire les outils de conciliation pour atteindre l'égalité recherchée. Enfin, le CESE a développé grâce à sa délégation à l'évaluation des politiques publiques et à la prospective un outil indispensable d'aide à la décision publique. Elle permet avec impartialité et pertinence de vérifier l'impact escompté et l'atteinte des objectifs qui étaient assignés à certaines politiques publiques. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter notre amendement.

permettre aux personnes tirées au sort de participer aux travaux des commissions du CESE, tout en préservant l'apport de Mme la rapporteure prévoyant que ces citoyens auront une voix consultative lorsqu'ils participent aux travaux des commissions du CESE. Cette disposition s'inscrit au coeur des avancées actuelles de notre société qui tendent à intégrer plus de démocratie participative dans le fonctionnement de nos institutions. Elle répond en cela aux aspirations de plus en plus fortes des Français. La démocratie participative a abouti ces dernières années à plusieurs succès. Lors du grand débat national, la question de la mise en place de procédures de tirage au sort des citoyens a été l'objet de nombreuses contributions en vue d'une meilleure association du citoyen à la prise de décision. Le tirage au sort a même fait l'objet d'une expérimentation s'agissant de la désignation des participants aux conférences citoyennes régionales, sortes de conférences locales organisées sous forme d'ateliers participatifs portant sur les différents thèmes du grand débat. De même, la Convention citoyenne pour le climat du Conseil économique, social et environnemental a été mise en place en octobre 2019 ; elle a réuni cent cinquante personnes toutes tirées au sort. Le recours au tirage au sort n'est pas nouveau dans notre démocratie, bien au contraire. On le connaît depuis bien longtemps, par exemple- sans rien confondre, madame la rapporteure ! -, pour la désignation des jurés d'assises. Pour autant, il ne s'agit aucunement ici de remettre en cause la démocratie représentative, qui demeure symbolisée par les deux assemblées parlementaires. Je vous invite donc à ne pas avoir peur du tirage au sort, à ne pas le dénigrer. C'est un outil de démocratie participative ancien, répandu à l'étranger dans de grandes démocraties, et qui n'a aucunement vocation à remettre en cause l'exercice du droit de vote.

les arguments que j'ai soulevés au titre de l'article 4 et fais mienne la démonstration de M. le garde des sceaux à l'instant.

qu'il me semble utile que le CESE puisse disposer de cet outil pour enrichir son travail par le biais d'une consultation sur un sujet donné.

pour explication de vote. Nous partageons la philosophie qui vient d'être décrite par notre collègue Leconte. Introduire le tirage au sort dans les travaux du CESE, c'est introduire

d'autre part, le côté « guichet unique de la concertation ». Ces deux points, même insuffisamment, ont été pris en compte par la commission des lois. Il reste néanmoins un manque manifeste sur la question de la démocratie participative.

marbre, même approximativement, des pratiques qui existaient déjà, nous sommes satisfaits d'avoir évité la procédure de tirage au sort, qui ne correspond pas à la conception que nous nous faisons de la participation des citoyens à la démocratie. Néanmoins, ce débat a permis d'échanger sur des sujets de fond, avec des désaccords de fond, aussi, avec un certain nombre de collègues. Je les remercie, en tant que rapporteur, de leur présence, de leur participation

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du